les réserves d'usage. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

l'État, en application de l'article L.741-2 du code de la construction et de l'habitation et de l'article L.321-1-1 du code de l'urbanisme. Or les périmètres d'intervention des EPF d'État ne couvrent pas l'ensemble du territoire national. Il est donc nécessaire de prévoir la possibilité d'intervention d'un autre opérateur, désigné par l'État, dans le cas où la commune où la commune dans laquelle est située l'ORCOD d'intérêt national n'est pas couverte par un EPF d'État. Cet amendement institue par ailleurs la possibilité, dans une ORCOD de droit commun, de déléguer le droit de préemption urbain à l'opérateur en charge de la conduite de l'ORCOD.

La loi du 10 juillet 1965 sur l'organisation et le fonctionnement des copropriétés ne prévoit aucune sanction à l'égard du syndic professionnel qui manquerait à ses obligations vis-à-vis du conseil syndical ou des copropriétaires. Le syndic étant le seul représentant légal du syndicat des copropriétaires, il ne peut s'assigner lui-même en cas de carence.

face aux carences du syndic. Il serait souhaitable de rééquilibrer les relations entre le syndic, le conseil syndical et les copropriétaires. Il faut également redynamiser les copropriétés pour répondre, par exemple, aux enjeux de rénovation des copropriétés, y compris de rénovation énergétique. Cet amendement prévoit

des situations, le syndic vous répond : « Vous avez certainement raison sur le fond, cher ami, mais, comme aucune sanction n'est prévue, je fais ce que je veux

je ne suis pas certaine qu'elle soit véritablement recevable sur le plan juridique, car cela permettrait à des copropriétaires de se faire en partie justice eux-mêmes.

toutefois tellement conscient de la difficulté que, dans le cadre des discussions que nous menons actuellement avec la Chancellerie pour modifier le texte,

peu probable que le syndicat des copropriétaires souhaite poursuivre sa collaboration avec lui. Sa révocation par l'assemblée générale paraît alors incontournable. Pour autant, confier cette action spécifiquement au président du conseil syndical nous semble soulever plusieurs difficultés. Outre qu'une telle disposition serait de nature à remettre en cause les grands équilibres de la gouvernance des copropriétés, elle conduirait également à accroître

Le président du conseil syndical n'a pas la personnalité juridique lui permettant d'ester en justice. Qui peut le faire ? Le syndic ! On demande donc au syndic de porter

ou administratives précises prévoient la levée du secret bancaire. Un tel amendement repose, en revanche, sur le souhait de particuliers que des problèmes rencontrés dans le cadre de leurs relations avec le syndic

Comment vérifier que celui-ci est bien habilité pour ce faire et qu'il n'agit pas à titre personnel ? Comment procéder aux vérifications imposées par les réglementations sur la lutte contre le terrorisme, qui prennent de plus en plus de place dans le travail quotidien des conseillers

par la voix du conseil syndical, ne peuvent se voir opposer le secret bancaire de l'article L. 511-33 du code monétaire et financier. Dont acte ! Monsieur

Cet amendement part du constat que la vente de logements sociaux entraîne, de fait, la création d'une copropriété. Si le bailleur assure généralement les fonctions de syndic, il a tout à fait le droit d'externaliser cette mission. Dans le même temps, il est aussi très fréquent qu'un tissu associatif existe dans ces immeubles et qu'il perdure après les opérations d'accession à la propriété. Dans ce cadre, la loi du 23 décembre 1986 précise que les représentants des locataires sont « invités » par le syndic à participer à l'assemblée générale et peuvent y prendre la parole sur tous les points inscrits à l'ordre du jour. Toutefois, vous en conviendrez, il s'agit d'une simple invitation, et non d'une convocation au sens strict, comme cela est prévu pour un copropriétaire. Autrement dit, le représentant des locataires ne se voit pas communiquer les différents documents venant en appui des résolutions prévues prévues à l'ordre du jour : arrêté des comptes, projets de contrats, devis ... De même, l'information peut lui être communiquée quelques jours seulement avant la tenue de l'assemblée générale, alors que les copropriétaires doivent être convoqués avec un délai de prévenance d'au moins trois semaines.

de la commission ? Actuellement, le syndic informe les représentants des associations de locataires, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de la date, de l'heure, du lieu et de l'ordre du jour de l'assemblée générale. Il s'agit d'une simple invitation

Le moins que l'on puisse dire est que la question des copropriétés semble, dans le cadre de ce débat, trouver enfin la place qui lui revient. Dans les problématiques du logement, on avait presque oublié que cette forme d'immeuble collectif fait largement partie du paysage urbain et que la centaine de milliers de copropriétés en difficulté polarise une bonne partie de la crise actuelle.

Selon une enquête de l'INSEE datant de 2013, un quart des copropriétés connaissent des situations plus ou moins avérées d'impayés de charges communes, pouvant conduire, comme on a pu le voir dans certaines situations déjà évoquées, à l'émergence, dans de très grands ensembles en difficulté, Il convient également de remarquer qu'un tiers des logements en copropriété sont occupés par des locataires et qu'un cinquième de ces logements ont acquis, avec le temps, le statut de résidence secondaire ou de logement vacant. La vacance de logements dans les copropriétés représentait, selon l'enquête de l'INSEE, l'équivalent d'un million de logements sociaux. Quand on cherche des solutions socialement acceptables au problème du logement, on pourrait se demander si la location à un niveau de loyer proche des plafonds sociaux de logements vacants dans des copropriétés ne pourrait constituer une voie à explorer. Cela étant, la présence plus ou moins importante de locataires en titre dans les copropriétés justifie, à notre avis, que ceux-ci soient pleinement informés de la vie de la structure et puissent notamment participer, dans les limites posées par leur situation, aux assemblées générales de copropriétaires régulièrement convoquées. L'article 44 de la loi Méhaignerie, qui entendait développer l'accession à la propriété par la revente de logements sociaux, entre autres démarches, avait reconnu aux associations de locataires représentatives un embryon de droits, que nous souhaitons ici renforcer, en faisant de la présence aux assemblées générales des représentants des locataires occupants une obligation.

Cette difficulté empêche de mettre en oeuvre des outils de gestion de ces espaces indivis, qu'il s'agisse de la nomination d'un syndic, de l'entretien et des travaux divers qui sont à réaliser. Des projets de rénovation en coeur d'îlot ne peuvent donc aboutir, et ce malgré la mise en place par les collectivités de dispositifs incitatifs auprès des copropriétaires. Ces cours communes non entretenues et ouvertes sur les voies publiques des centres-villes entraînent une dégradation de la qualité des espaces collectifs, ainsi qu'une baisse de l'attractivité des logements.